L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les directeurs d'école sont un rouage essentiel au bon fonctionnement de nos écoles primaires. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des familles, des élus locaux ou de l'autorité hiérarchique. La proposition de loi de notre collègue députée Cécile Rilhac apporte un fondement juridique à leur action et à leurs missions, qui sont toujours plus nombreuses. Elle s'inscrit dans une dynamique née d'une volonté partagée par le Parlement et par le Gouvernement d'améliorer la situation des directeurs d'école. d'école. Le ministre de l'éducation nationale a d'ailleurs pris récemment plusieurs mesures en ce sens. Le texte que nous examinons aujourd'hui a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire le 16 novembre dernier. Je tiens à saluer le travail de notre rapporteur, Julien Bargeton, qui a travaillé de concert avec Max Brisson, Sonia de La Provôté, notre collègue députée Cécile Rilhac et les présidents des commissions de la culture de nos deux assemblées pour aboutir à ce texte d'équilibre. Cette proposition de loi constitue une occasion importante en faveur de la reconnaissance du rôle des directeurs d'école. Surtout, elle a vocation à faciliter la vie de l'école au quotidien. Elle rend possible la délégation de compétences de l'inspecteur de l'éducation nationale au directeur d'école, dans la perspective d'une gestion de proximité adaptée aux caractéristiques propres à chaque école. Par ailleurs, et c'est un apport majeur du Sénat, le directeur d'école se voit reconnaître une autorité fonctionnelle pour le bon fonctionnement de son école. Les directeurs d'école veulent du temps, une formation et des moyens. Ce texte reconnaît pour la première fois dans la loi le principe du temps de décharge. Nous avons souhaité que ce temps soit suffisant pour permettre aux directeurs d'accomplir l'ensemble de leurs missions

le recteur, ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, devra présenter chaque année un bilan de l'utilisation des décharges et de leurs motifs- nous avons tenu à ce que cette disposition introduite par le Sénat

La proposition de loi permet également de décharger les directeurs d'école d'un certain nombre de tâches ; je pense à l'élaboration du plan de sécurité de l'école. La consultation lancée voilà deux ans par le ministère de l'éducation nationale auprès des directeurs d'école montre qu'il s'agit d'une mission jugée pénible,

En outre, le directeur d'école ne participera plus aux activités pédagogiques complémentaires, sauf s'il est volontaire. Sur l'initiative du Sénat, nous renforçons la formation des directeurs d'école, dès le stade de la formation initiale des futurs enseignants, mais aussi avant leur prise de poste en tant que directeur, puis tout au long de leur carrière. Ce texte prévoit également la mise en place dans chaque département d'un référent direction d'école dont le rôle est d'épauler les directeurs et de répondre à leurs questions, avec un objectif : faire en sorte qu'ils ne se sentent plus seuls. Enfin, les directeurs d'école veulent des moyens ; il était inenvisageable de faire abstraction de cette demande. À cet égard, l'article 2 traduit la satisfaction de notre objectif partagé, à savoir la reconnaissance des moyens dont les directeurs et directrices ont besoin. le sais, cet article est celui qui a été le plus débattu, y compris au sein de notre assemblée, mais il serait paradoxal qu'un texte consacré aux moyens des directeurs d'école n'évoque pas les communes et leurs groupements. Les collectivités locales constituent, après l'État, le premier financeur des dépenses d'éducation. Dans le premier degré, les communes et leurs groupements y participent à hauteur de 33 %. Cette contribution financière est essentielle au bon fonctionnement de nos écoles primaires. La rédaction de l'article 2 issue de la commission mixte paritaire évite tout risque de transfert de charges entre l'État et les collectivités locales.

Les communes ont la charge de l'entretien et du fonctionnement de l'école, c'est-à-dire de l'aide matérielle. Cette proposition de loi s'est enrichie et améliorée au fil des deux lectures. Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire reprend un grand nombre d'apports du Sénat. L'empreinte de notre assemblée y est forte.

Je le sais parce qu'il me l'a dit, il aurait été très heureux d'être parmi vous pour ce moment important, car il a fallu du temps pour que ce texte trouve son point d'équilibre. Malheureusement, il est retenu par une réunion avec le Premier ministre sur la situation sanitaire,

... Durant la pandémie, matin et soir, les directeurs et directrices d'école ont continué de faire face en organisant en toutes circonstances la continuité des enseignements. Si notre

au quotidien. Elle s'inscrit dans la droite ligne de ce que nous avons fait jusqu'ici et porte l'ambition de conforter et de sécuriser l'emploi

le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte. En conséquence, le vote sur les articles sera réservé.

elles lui sont en réalité bien antérieures ; en témoignent les démissions au sein du corps enseignant, de plus en plus nombreuses chaque année. Les directeurs et directrices d'école comptent au nombre des figures de proue de cette institution ils et elles subissent donc fortement les secousses qui l'affectent, et sont confrontés, dans l'exercice de leurs missions, à des difficultés spécifiques. Ces difficultés, nous ne pouvons feindre de les ignorer, car elles sont connues de longue date

Certes, cette proposition de loi comporte quelques avancées, et je tiens en la matière à souligner l'apport de la chambre haute, qui a notamment permis l'instauration d'un point annuel sur l'effectivité de l'utilisation des décharges

les décharges et l'aide administrative et matérielle apportée aux directeurs et aux directrices. Sur ce deuxième point, la déception est d'autant plus grande que le Sénat s'était prononcé, à plusieurs reprises, à l'occasion des différentes lectures, en faveur d'une formule claire, consacrant les responsabilités de l'État en la matière. Nous, membres de la chambre des territoires, savions qu'il serait peu judicieux de charger les collectivités de nouvelles prérogatives. Imaginez donc notre surprise, de la commission mixte paritaire, quand nous avons découvert que la formulation retenue mentionne de nouveau aussi bien l'État que les collectivités, et ne fixe d'obligation pour aucun de ces acteurs. Nous voilà presque revenus à la rédaction de l'Assemblée nationale, dont les travers avaient pourtant été dénoncés avec force sur toutes les travées de notre hémicycle Ne nous y trompons pas, l'article 2 tel qu'il est formulé aujourd'hui, témoignant d'un refus de trancher, ne résout strictement rien. La version finale du texte persiste, par ailleurs, à élargir le champ des missions des directeurs et directrices en leur confiant un rôle de formation, alors même que le constat de leur surcharge de travail était unanimement partagé par toutes et par tous. Enfin et surtout, une ligne franchie l'introduction d'une notion mal définie, celle de l'autorité fonctionnelle, qui s'est imposée malgré nous, au fil de nos débats, comme la bonne réponse au mal-être éprouvé par les directrices et les directeurs. S'il nous a été dit et répété que cette autorité fonctionnelle n'était pas synonyme d'autorité hiérarchique, l'ambiguïté demeure en raison, en particulier, du refus d'énoncer clairement cette précision dans le texte. Cette évolution, introduite par la majorité sénatoriale avec le soutien du pouvoir exécutif, est d'autant plus surprenante qu'elle va à rebours des attentes des directeurs et directrices, qui souhaitent avant tout être soulagés de façon très très concrète dans l'exercice de leurs missions, et non assumer un rôle d'autorité auprès de leurs pairs enseignants. Elle fragilise le fonctionnement collectif de l'école primaire républicaine tel qu'il fut imaginé par Jules Ferry, dont la clef de voûte était jusqu'à présent le conseil des maîtres. Cette notion d'autorité fonctionnelle résonne de façon d'autant plus inquiétante qu'en septembre dernier, à Marseille, le Président de la République nous exposait sa vision libérale de l'école et du rôle des directeurs et directrices, clairement inspirée du monde de l'entreprise et à mille lieues de notre conception de l'école républicaine, indissociable de la fonction publique. Vous l'aurez compris, notre groupe ne votera pas en faveur de cette proposition.

Je félicite de nouveau Cécile Rilhac, notre collègue députée, comme je l'avais fait en première lecture, pour avoir été à l'initiative de ce texte, pour l'avoir défendu avec conviction et accompagné jusqu'au bout. Une fois adoptées, ces mesures dont nous discutons rendront possibles des avancées significatives en faveur des directrices et directeurs d'école. Elles amélioreront la reconnaissance de leur rôle. Elles fixeront un cadre juridique bienvenu, permettant de conforter leur légitimité et leurs actions.

permettra aux directrices et aux directeurs d'assurer le bon fonctionnement de leur école en renforçant leur pouvoir d'initiative et de décision. Je le précise, car en la matière la caricature est toujours possible : il s'agit d'une autorité fonctionnelle et non hiérarchique. Demain, grâce à une meilleure articulation des missions, les temps de décharge seront plus effectifs. En effet, le texte prévoit que ces indispensables décharges soient déterminées en fonction du nombre de classes et des spécificités de l'école. Demain, un cadre juridique spécifique explicitera les conditions applicables à la nomination des directrices et directeurs d'école, ainsi qu'à leur formation et à l'exercice de leur fonction.

L'État et les communes restent chacun dans leur champ de compétences respectif : les communes et leurs groupements peuvent mettre des moyens matériels à disposition des directeurs d'école, tandis que l'État peut leur fournir une assistance administrative. Cette rédaction n'impliquera donc pas de transfert de charges de l'État vers le bloc communal ; nous pouvons nous en féliciter. Pour toutes ces raisons, notre groupe, qui s'était abstenu en seconde lecture, votera ce texte. En conclusion, je voudrais évoquer le budget de l'éducation nationale. Premier poste dans le projet de loi de finances pour 2022, à 56,5 milliards d'euros, soit une hausse de 1,7 milliard d'euros. Cette augmentation inclut notamment les près de 700 millions d'euros promis voilà quelques mois par Jean-Michel Blanquer pour revaloriser les salaires des enseignants.

Je salue le travail réalisé lors des lectures successives par les deux assemblées à partir de l'initiative de Mme Cécile Rilhac. Nos travaux ont été largement documentés par les conclusions du rapport d'information sénatorial sur la situation des directeurs d'école. La reconnaissance et la valorisation de leurs fonctions au travers d'un cadre juridique clair figurent au centre des préoccupations que nous partageons.

Ces modalités sont indispensables pour permettre à de nombreuses écoles en milieu rural de disposer d'un enseignant faisant fonction de directeur ; loin d'être anecdotique, cette situation concerne une école sur quatre. Fidèles à la vocation du Sénat, nous avons également veillé à préserver une juste complémentarité des compétences entre État et collectivités. la commission mixte paritaire est parvenue à un équilibre permettant de renforcer les moyens mis à disposition des directeurs d'école sans alourdir les charges qui pèsent sur les communes et les intercommunalités. La commune pourra mettre à disposition des directeurs des moyens matériels, tandis que l'État garantira la mise à disposition d'une assistance administrative, dans le cadre de la politique éducative menée par le Gouvernement. La suppression par le Sénat de l'article 4 sur le temps périscolaire a été maintenue à l'Assemblée nationale. La proposition consistant à associer le directeur d'école à l'organisation du temps périscolaire est pourtant intéressante. Je rappelle qu'il s'agissait bien d'une possibilité, encadrée par un dispositif juridique adapté et souple, et non d'une obligation. L'association du directeur d'école à l'organisation du temps périscolaire aurait permis d'instaurer un continuum dans la prise en charge des enfants. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires y était favorable, à condition de prévoir les temps de décharge nécessaires. Je souhaite attirer votre attention sur le rôle central des directeurs d'école en matière de climat scolaire et de lutte contre le harcèlement. J'ai eu l'honneur d'échanger hier avec Mme Brigitte Macron, très impliquée sur ce sujet, dans le cadre d'un entretien que nous avons eu à la suite de la publication du rapport de la mission d'information sénatoriale Nous avons évoqué notamment l'importance de mobiliser dès l'école élémentaire l'ensemble des enseignants, le directeur, autour de l'apprentissage des droits et des devoirs des élèves et de la juste valeur des mots, ainsi que de l'application pratique du droit à une scolarité sans harcèlement consacré par la loi pour une école de la confiance. Les directeurs d'établissement sont des acteurs indispensables de la lutte contre la violence à l'école. En effet, ils sont amenés à participer de façon active à la prévention, à la détection et au suivi des situations de harcèlement, pour permettre à chaque enfant de bénéficier d'une scolarité sans violence et prévenir les drames. Pour toutes ces raisons, cette proposition de loi est particulièrement attendue par l'ensemble de la communauté éducative. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire.

nous voici réunis pour l'ultime examen de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école. Après de longues heures de discussion et un intense parcours législatif, l'accord entre les deux assemblées est désormais possible. Je m'en réjouis.

Je crois pouvoir ajouter que la rédaction proposée est juste et équilibrée. Elle matérialise la volonté commune de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Gouvernement d'améliorer significativement la situation des directeurs d'école. Aussi, je souhaite saluer le travail de notre rapporteur Julien Bargeton ainsi que, bien entendu, celui de Cécile Rilhac, auteure de cette proposition de loi. Avec l'un comme avec l'autre, ainsi qu'avec Sonia de La Provôté, nous avons pu agir en profondeur- et en toute confiance. Je les en remercie. Noyau dur de cette proposition de loi, l'autorité fonctionnelle est octroyée. Les mots ont été choisis, pesés et posés : ce sont ceux du Sénat. Contrepartie de responsabilités accrues, les directeurs auront désormais, pour les assumer, l'autorité sur les professeurs de l'école qu'ils dirigent. Ils participeront à l'encadrement et à l'organisation de l'enseignement du premier degré. C'est une réelle rupture

La rédaction actuelle du texte, sur laquelle nous nous sommes accordés, répond au moins partiellement à ces besoins. Et le Sénat a été le principal moteur des avancées qu'il contient. Ainsi, nous avons fixé un cadre précis,

Si les deux assemblées s'accordaient sur le caractère nécessaire de la mesure, il n'y avait pas de consensus quant à savoir à qui devait incomber cette charge. Pour le Sénat, il n'était pas envisageable que les communes et leurs groupements en soient responsables. Nous nous y sommes fermement opposés.

à l'État, mais celui-ci n'impose rien non plus aux collectivités locales. Voilà ce que le Sénat a obtenu ! En revanche, État et collectivités peuvent répondre à une demande qui s'avère en particulier pressante dans les écoles de moyenne et de grande taille. Le texte que nous allons adopter aujourd'hui est donc le fruit d'intenses échanges. Nous avons réussi à trouver une rédaction consensuelle ; d'une importance capitale pour l'exercice de la fonction de directeur d'école, elle évite de surcroît des effets de bord qui auraient pu être lourds de conséquences pour les collectivités. « Un chef, c'est fait pour cheffer », affirmait le président Jacques Chirac. Par ce texte, nous avons enfin donné corps à l'emploi de directeur d'école et assorti cette fonction

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous arrivons aujourd'hui au terme de la discussion de ce texte, qui était très attendu par les directrices et directeurs d'école.

Le texte apporte quelques réponses au sujet des décharges de classe, du moins en théorie. Mais ces mesures seront-elles suivies d'effet dans la pratique ? Nous pouvons en douter, eu égard aux difficultés de recrutement ou de remplacement déjà constatées dans certaines académies.

Les directrices et directeurs d'école manquent de temps et leurs tâches se multiplient. Le texte devait répondre à cette surcharge de travail, au lieu de quoi il leur est demandé d'accomplir des tâches supplémentaires, comme celle de proposer des actions de formation. Allons-nous dans le bon sens ?

Il aurait été plus fort de conserver la formulation proposée par le Sénat ; de réelles avancées auraient suivi. Évidemment, il aurait aussi fallu aller plus loin en exigeant que cette aide administrative

bout du compte, on peut craindre que ce texte ne soit que la première marche vers la concrétisation d'une vision managériale de l'école promue par le Président de la République. La prochaine étape sera-t-elle de transformer les directrices et directeurs d'école en chefs d'entreprise recruteurs ?

Les directeurs d'école demandent plutôt une revalorisation de leur fonction. On entend gérer la pénurie de postes en assouplissant les conditions d'accès à la fonction de directeur- termes, on s'attaque aux conséquences plutôt qu'aux causes. Mais casser le thermomètre n'a jamais fait baisser la fièvre, j'en parle en connaissance de cause ! Une nouvelle architecture se dessine ainsi. n'est pas certain que la réussite des élèves et la réduction des inégalités, qui restent les principaux enjeux de l'école, aient à y gagner. Si je suis revenue, au début de mon propos, sur l'histoire de cette volonté de modifier le statut des directeurs d'école,

carte. Je me félicite que la CMP n'ait pas retenu l'inscription des formations dans le cadre des orientations nationales. Mieux, elle lui a substitué un renforcement du rôle du conseil des maîtres,

des travaux de cette CMP : la suppression des formations certifiantes, dont les contours nous semblaient bien trop flous, et le maintien d'un rapport annuel sur l'effectivité des décharges et des remplacements- chacun sait que le problème du remplacement est un problème structurel et que les décharges

lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient. En l'état, cette assistance administrative risque de demeurer un voeu pieux alors même qu'elle est la demande essentielle que formulent les directeurs Notre école a besoin de directeurs dont les tâches administratives sont allégées par l'octroi d'un temps de décharge ou d'une aide suffisante, afin qu'ils puissent se recentrer sur la coordination et l'animation des équipes pédagogiques. Je crains que le concert de satisfaction que j'entends ici

quelle que soit la taille de l'école, est un bon compromis. Elle permet une formation tout en évitant l'écueil de la raréfaction des candidats, qui est une réalité sur le terrain. Quant à l'obligation d'offrir une formation continue aux directeurs d'école,

Cette clarification du rôle de chacun était indispensable. Madame la secrétaire d'État, mes collègues du groupe Union Centriste et moi-même saluons ces dernières dispositions confirmées, clarifiées, améliorées. Nous nous réjouissons tous de l'esprit de ce texte utile, attendu, qui consacre le rôle des directrices et directeurs d'école au sein de l'éducation nationale et sera un véritable outil à leur service au quotidien. Être directeur ou directrice d'école est un engagement. Cette mission ne doit pas être une obligation. Elle est avant tout un choix au bénéfice des enfants et de l'éducation. L'adoption de ce texte constitue ainsi une reconnaissance de ces véritables piliers de l'école de la République, qui en sont les garants, tous les jours, dans tous les territoires.